Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, fer de lance de la politique d’accès des jeunes à la culture depuis sa création en 2019 et sa généralisation en 2021, le pass Culture

posé ce diagnostic en demi teinte : les résultats du pass Culture sont jugés satisfaisants sur un plan quantitatif, mais insuffisants pour diversifier les pratiques culturelles des utilisateurs. Un an plus tard, l’inspection générale des affaires culturelles dressait un constat similaire, mettant à son tour en doute la capacité du pass Culture à atteindre ses objectifs de service public. En décembre dernier, la Cour des comptes a étayé ce constat et confirmé les nombreuses limites du dispositif, en insistant sur son dérapage budgétaire.

peu compatible avec les objectifs de démocratisation et de diversification culturelles. Jean Raymond Hugonet, chargé dès 2018 d’animer un groupe de suivi à ce sujet,

au détriment d’autres actions, comme l’éducation artistique et culturelle (EAC), à laquelle nous sommes tous, sur ces travées, particulièrement attachés. Le pass Culture semble donc avoir échoué à être le sésame de la démocratisation et de la diversification des pratiques culturelles des jeunes. Sa suppression pure et simple, évoquée par certains, serait toutefois irréaliste et surtout préjudiciable à nombre de secteurs culturels. Tout d’abord, l’outil est désormais mis en œuvre et plébiscité : 94 % des jeunes s’en sont saisis. Ceux qui ont été auditionnés à l’occasion d’une table ronde dédiée au pass Culture dans le cadre de nos travaux budgétaires ont souligné combien ils appréciaient l’autonomie et la liberté de choix que ce dispositif leur offrait. Cette poche de liberté permet à certains d’entre

ont vu des jeunes franchir pour la première fois leur porte, écouter leurs conseils de lecture et revenir une fois le pass utilisé.

collectivement aux modalités d’un recalibrage à la fois stratégique et budgétaire du pass Culture. Quels contours cette réforme pourrait elle prendre ? Le principe de libre choix des jeunes, qui constitue l’essence même du volet individuel du

ne garantit pas, à elle seule, la diversification des pratiques. Sans accompagnement spécifique à même de susciter leur curiosité, les jeunes pourraient ne pas s’en saisir. Les montants de la part individuelle

le montant soit modulé en fonction des ressources. Cette piste nous semble intéressante, même si elle présente certaines difficultés techniques de mise en œuvre. Peut être pourrez vous nous dire, cette après midi, comment vos services ont avancé sur ce sujet. Cette mise sous condition de ressources ne suffira bien sûr pas à combattre les inégalités sociales d’accès à la culture. Là encore, des mesures d’accompagnement par les tiers seront incontournables. C’est pourquoi les membres de notre commission vous le disent avec force : le développement de la médiation culturelle est un préalable indispensable à toute réforme du pass Culture. Nous attendons donc, de votre part, des garanties sur ce volet jusqu’ici trop négligé. Un autre sujet nous préoccupe : l’accès aux infrastructures culturelles pour les jeunes qui en sont éloignés, notamment dans les territoires ruraux. La prise en charge des frais de transport fait elle partie des options retenues, à ce titre, engager un dialogue avec les collectivités territoriales ? Par ailleurs, le continuum entre la part individuelle et la part collective doit être retravaillé, car celles ci se

culturelles (Drac) la possibilité de soutenir des initiatives culturelles décloisonnées et adaptées au contexte des différents territoires. Ce fonds visait à répondre à une proposition émise par Sonia de La Provôté et Sylvie Robert dans leur

: le soutien à la création, à l’éducation artistique et culturelle et aux établissements d’enseignement passe par un dialogue approfondi entre État et collectivités territoriales, ainsi que par le développement de nouvelles modalités de contractualisation.

les jeunes consacrent d’ailleurs une part plus importante de leur pass à l’offre numérique. Les élus du groupe écologiste reconnaissent que le pass Culture fait désormais partie du paysage culturel et que sa suppression serait mal comprise, notamment par les enseignants, qui en font un usage formidable.

comme règle de droit, en omettant trop souvent les attentes réelles du public ? Est ce vraiment leur rôle d’exposer de la sorte le pass Culture à des polémiques qui dégradent l’image d’une initiative pourtant appréciée des Français ? Lors du débat budgétaire, vous avez déclaré vouloir réorganiser ce comité et son mode de fonctionnement. Vous venez de nous indiquer les voies de transformation

Madame la ministre, vous avez annoncé vouloir que les usagers du pass se tournent davantage vers les libraires indépendants, la presse écrite et le spectacle vivant,

Surtout, on constate que le coût de la part individuelle du pass est systématiquement supérieur aux dotations initiales. Selon la Cour des comptes, des arbitrages doivent être pris afin de mettre un terme à cette croissance non maîtrisée des dépenses. La Cour a présenté trois pistes d’économies réduire le montant du crédit alloué aux jeunes de 18 ans ; le soumettre à des conditions de ressources ; et cibler les bénéficiaires selon des critères sociaux ou territoriaux. Par ailleurs, il semble souhaitable de transformer la SAS en opérateur public afin qu’un contrôle plus étroit de son action puisse être exercé par le ministère et par le Parlement.

La part collective donne satisfaction et mérite d’être développée, même si des évolutions sont nécessaires. Les enseignants se sont approprié l’outil : le pass leur donne les moyens de prendre des initiatives et nourrit incontestablement l’éducation artistique et culturelle dans les établissements.

ce dispositif peine à être un outil d’émancipation culturelle et d’accès à la culture pour ceux qui en sont le plus éloignés ». La part individuelle du pass Culture coûte à l’État près de 250 millions d’euros par an, soit le triple de la part collective, dont j’ai souligné à la fois l’intérêt et le potentiel. Dès lors, on s’interroge…

Il doit donc encore faire ses preuves en tant qu’outil de démocratisation de la culture. Certes, il s’est déjà progressivement ajusté. À preuve, 84 % des jeunes sont inscrits ; mais en bénéficient ils ? C’est une autre affaire… Le livre reste le plus présent dans les dépenses, et la part des mangas a été divisée par deux en trois ans. Le récent recours à la médiation culturelle a renforcé l’utilisation du pass Culture en faveur du spectacle vivant, dont la fréquentation a augmenté de 30 % en quelques mois.

une SAS publique était une solution quelque peu incongrue et difficile à suivre… En effet, des zones d’ombre demeurent. L’équation financière du pass reste nébuleuse et son fonctionnement particulièrement intrigant. De plus, il devait, au départ, être financé à hauteur de 80 % par des ressources extérieures.

Dans la discussion générale, la parole est à Mme Nathalie Goulet, auteur de la proposition de loi. Madame Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il est assez rare qu’un texte somme toute peu ambitieux fasse ainsi l’unanimité contre lui

Madame la présidente, monsieur le ministre,

le Sénat a eu à cœur de mener un travail de simplification des normes et des procédures, au service des citoyens et des entreprises. La maîtrise du nombre de ces instances en fait pleinement partie.

de facilité pour le Gouvernement et pour le législateur. La réduction de leur nombre tend à marquer le pas ; celui ci a même augmenté en 2022 et en 2023, et l’année 2024 n’a vu la suppression nette que d’une seule instance.

devenues caduques ou inutiles. Avant d’entrer dans le détail du texte, permettez moi de souligner que, si l’objet de cette proposition de loi est vaste, les instances délibératives et consultatives qui y sont mentionnées sont, en matière de simplification administrative, l’arbre qui cache la forêt. Le nombre, le coût et les prérogatives confiées à ces instances sont sans commune mesure avec ceux des opérateurs et des agences de l’État. L’enchevêtrement des compétences, les coûts pour les finances publiques et la lenteur administrative provoqués par ces derniers

Je me réjouis donc de la décision, prise hier par la conférence des présidents, de créer une commission d’enquête sénatoriale sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l’État, afin de dresser un constat complet et objectif de l’utilité de toutes ces instances.

leur création, parfois très récemment. Eh oui ! Veillons donc à ne pas légiférer à la hâte, à ne pas supprimer des instances qui permettent au Parlement d’exercer ses missions de suivi et de contrôle de l’action gouvernementale. Au reste, d’autres structures ont été créées pour favoriser le dialogue et la concertation

En conséquence, la suppression de quatre instances a été écartée lors de l’examen en commission. Il est en effet apparu qu’elles assuraient un éclairage utile tant au Gouvernement

De Gaulle disait : « L’essentiel […], ce n’est pas ce que peuvent penser le comité Gustave, le comité Théodule ou le comité Hippolyte ; l’essentiel […], c’est ce qui est utile au peuple français, ce que sent, ce que veut le peuple français.

cette contribution à la lutte contre le fameux « millefeuille administratif » de notre pays s’inscrit dans un cadre plus vaste, celui de la simplification, chantier que j’entends conduire en tant que ministre.

Nous le savons tous, l’effort de suppression de ces comités ne contribue pas significativement à l’effort d’économies budgétaire – il faut être lucide. Toutefois, ce travail concourt à une meilleure lisibilité de l’action publique. C’est la dimension symbolique de la simplification. Cette proposition de loi est importante, car elle viendra nourrir les réflexions de l’Assemblée nationale sur l’article 1 du projet de loi de simplification de la vie économique.

À ce titre, je soutiens son initiative de lancer une commission d’enquête sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l’État, laquelle permettra d’évaluer finement leurs coûts et leurs missions. Je suivrai avec attention ces travaux, qui contribueront à alimenter notre réflexion pour réformer en profondeur l’organisation de l’État. Comme vous le savez, M. le Premier ministre a annoncé très clairement sa volonté de réformer l’organisation de l’État et de rationaliser l’action de ses agences. Cette décision s’inscrit dans un effort au long cours : je ne peux pas vous laisser dire que l’État n’a pas agi ces dernières années en la matière. Depuis 2010,

Évidemment, si je voulais être populaire, je vous promettrais du sang, des larmes et des coups de tronçonneuse. Mais je ne suis pas de ceux qui adoptent des postures radicales à des fins de communication. Au contraire, je suis convaincu que nous devons aborder cette question de manière pragmatique,

Disons le : quand on rase une forêt au bulldozer, on abat aussi des arbres en bonne santé, dont la présence est essentielle. Oui, je suis convaincu que nous devons simplifier. Oui, je crois que c’est vital pour l’efficacité de l’action publique. Non, je n’aurai pas la main qui tremble pour supprimer des comités, dès lors que nous aurons prouvé leur inefficience.

Enfin, changeons de regard sur la simplification. La charge de la preuve doit être inversée : au lieu de chercher à établir l’inutilité d’un comité, regardons d’abord ce qu’il apporte à nos concitoyens. Sortons de la critique facile au profit d’une analyse objective : c’est ce que nos concitoyens attendent de nous. Mesdames, messieurs

singulièrement l’ambition de ce texte. Certains articles suscitent toujours des interrogations, car ils visent à abolir des structures dont le travail est reconnu,

À ceux qui réclament toujours plus d’argent public et qui répètent que l’État n’en fait jamais assez, il faut répondre que le périmètre de ce dernier est trop étendu : à vouloir trop faire, il fait mal ! Cette suractivité étatique, observée lors de l’examen du budget, favorise aussi la prolifération de normes et comités. À ce titre, mon collègue des Ardennes, le maire de Charleville Mézières Boris Ravignon,

dans les législateurs deux penchants naturels, le besoin d’agir et le plaisir de se croire nécessaires ». Hélas ! Ce qui est vrai pour les lois l’est aussi pour les comités consultatifs. Évidemment, certains parmi ces derniers sont utiles et nous devons nous garder de les supprimer trop hâtivement. Sans une étude précise de leur fonctionnement et de leur activité réelle, nous ne pourrons pas traiter efficacement le problème. Une commission d’enquête sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l’État verra bientôt le jour. Nous sommes convaincus que les frais de fonctionnement, le nombre d’ETP ou encore les locaux que les agents occupent méritent d’être évalués par la représentation nationale.

plus de deux décennies, celle ci vise à amorcer concrètement la rationalisation administrative et la réduction des dépenses. Il s’agit là des prémices d’un long cheminement qui consistera non pas à tout faire disparaître, mais bien à évaluer, tous ensemble, l’efficience de telle ou telle structure, son utilité et la pertinence de maintenir son indépendance, de l’intégrer à son ministère de référence ou, tout simplement, de procéder à des suppressions afin d’éviter les superpositions d’expertises. exigence résulte de la mission de contrôle parlementaire que doit exercer le Sénat. Le document annexé au projet de loi de finances, dit jaune budgétaire, dresse la liste exhaustive des comités, conseils, commissions, observatoires et autres.

près de soixante autres conseils disposent de budgets parfois importants. Que dire également du secteur agricole, déjà saturé d’agences et d’opérateurs publics ? L’objectif n’est pas de remettre en question la bonne foi ou la compétence des personnes impliquées dans ces structures, bien qu’il soit parfois tentant d’examiner de plus près les liens entre les nommés et ceux qui les nomment… Il s’agit plutôt de rendre plus lisible l’action publique.

Monsieur le ministre, vous pourrez compter sur le Sénat dans les prochains mois pour scruter la moindre piste d’économies au sein de l’État ! Au delà du bien fondé de ces comités et de leur financement, il conviendrait aussi de s’interroger sur l’usage

de résultat plutôt que de moyens, en demandant aux organismes des propositions concrètes dans leur domaine de compétences. Par exemple, le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP) pourrait fournir des recommandations d’économies directement exploitables par le ministre de l’économie et des finances. Enfin, je tiens à souligner l’intérêt de procéder à un mouvement de rationalisation et de fusion plutôt qu’à des suppressions brutales. Je salue à cet instant le travail de la commission des lois et du rapporteur, Hervé Reynaud, lequel a su défendre une approche bienveillante afin de favoriser une gestion

tout du moins le vaccin permettant de nous immuniser contre l’inutilité ou le « doublonnage » des actions, à en faire pâlir les complotistes les plus aguerris ? vont dans le bon sens et constituent un premier pas vers la rationalisation des services de l’État, même s’il est nécessaire de pousser la réflexion bien au delà de la suppression d’une quinzaine d’instances, dont accouchera probablement ce texte. Gardons en tête que le besoin d’exister de certains de ces comités se concrétise parfois par l’art de complexifier le quotidien quotidien de l’État ou des collectivités ! Vous l’aurez compris, mes chers collègues, les membres du groupe Les Républicains sont plutôt favorables à cette proposition de loi. Ils ont d’ores et déjà fait savoir qu’ils souhaitaient aller plus loin en

Récemment, à l’occasion de sa déclaration de politique générale, l’ancien Premier ministre Gabriel Attal a proposé la règle suivante, que vous avez rappelée, madame Goulet : la suppression de « tous les organes,

non titulaire d’un diplôme français souhaite exercer la profession de conseiller en génétique sur notre sol. Cette structure tend à éclairer la décision du préfet de région sur la délivrance de cette habilitation à exercer. Face aux progrès thérapeutiques et à la recherche médicale, en particulier sur le génome humain dans le cadre des très lourdes pathologies, ne faudrait il pas conserver ce filtre d’expertise ?

Cette dernière se prononce sur toute question relative aux pratiques commerciales lui étant soumise, afin de contribuer à la résolution de conflits entre acteurs commerciaux dans un univers qui se complexifie. Elle assure également un travail de clarification normative à l’égard de l’ensemble des parties prenantes à la chaîne de production et de distribution, notamment en matière agricole. Il ne faudrait pas supprimer ce qui permet de simplifier

À titre liminaire, je tiens à affirmer l’attachement de l’ensemble du groupe RDSE à la maîtrise des dépenses et à la simplification de l’action publique.

Je remercie mes collègues Nathalie Goulet et Hervé Reynaud de leur travail. Leur investissement nous permet de débattre de ce sujet aujourd’hui. Surtout, cette discussion est un appel à l’humilité, car elle nous conduira sûrement à supprimer des instances dont le législateur est à l’origine. Je souligne d’ailleurs l’attachement tout particulier de Christian Bilhac à cette démarche, lui qui se bat contre le recours excessif aux agences dans la gestion publique. Bien que je ne souscrive pas personnellement aux amendements qu’il a déposés,

Bien que j’entende les arguments selon lesquels ces organes ont été sélectionnés selon des critères d’activité ou de chevauchement de compétences, il me semble que de telles décisions doivent faire l’objet d’une concertation plus complète pour garantir leur acceptabilité. ne doit pas être de nature à créer des tensions au sein des publics concernés. Je me satisfais toutefois que le travail du rapporteur ait permis d’identifier des instances qui méritent de perdurer. Un tel résultat doit justement nous appeler à la prudence.

ce texte me paraît une invitation pertinente à la discussion sur un sujet prégnant. Nous devons apporter une réponse à la hauteur de la situation budgétaire de notre pays et digne de l’appel de nos concitoyens à la simplification. Que nous adoptions les dispositions proposées ou non, j’appelle à ce que ce premier travail soit suivi d’une évaluation méticuleuse qui permettra d’identifier les conséquences de la suppression comme du maintien

cette proposition de loi est un test. En effet, mes chers collègues, elle représente un premier jalon ou un premier signal. Il s’agit de démontrer notre volonté de simplifier concrètement l’action publique en la rationalisant – et nous sommes attendus ! Ce texte, Ce texte, sur l’initiative de Nathalie Goulet, doit être le témoin de notre volonté de rendre l’administration plus efficace, plus lisible et mieux adaptée aux défis contemporains.

et dont la compétence dans le domaine est reconnue, telle que l’Agence nationale du sport. Nous formulons une proposition en ce sens. Nous avons conscience que la lisibilité de l’action publique conditionne directement la confiance que nos concitoyens placent dans nos institutions. Pour cette raison, maintenir ce type de commissions qui n’ont pas d’activité est simplement contre productif. Nous ajoutons de la complexité et de l’opacité là où l’État doit, au contraire, simplifier, rationaliser et clarifier. Il y va de la crédibilité de nos institutions Soyons honnêtes : cette prolifération est tout à fait déraisonnable et ne peut qu’attirer, à juste titre, des regards circonspects, voire ironiques, ne serait ce qu’en raison de l’intitulé de certains de ces « hauts » comités… En simplifiant le paysage administratif, nous démontrerons que l’État est capable de se remettre en question et de faire le tri entre ce qui est nécessaire et ce qui ne l’est pas. Même si la méthode doit être affinée,

aucun d’entre nous n’aurait l’idée de cotiser à un organisme qui ne se réunit pas ou de s’abonner à une revue qui ne publie rien ! Nous ne trouverons pas là de miraculeuses économies

En actant par son adoption notre volonté de supprimer des structures devenues obsolètes qui mobilisent encore des ressources, même modestes, et qui ralentissent les processus décisionnels,

Je salue le travail de la commission des lois et de son rapporteur, M. Hervé Reynaud. Cependant, faisant écho aux propos tenus précédemment par Nathalie Goulet, je suis tout de même réservée quant au raisonnement privilégiant la « démonstration de l’inutilité » d’une structure pour accepter sa suppression plutôt que la preuve de son utilité pour justifier son maintien. J’en profite, ici, pour faire un clin d’œil à mon collègue élu depuis moins longtemps que moi, et lui dire que Nathalie Goulet a souvent le tort d’avoir raison avant tout le monde ! Je me souviens d’un texte, également martyr, dont elle fut l’auteur en 2020, appliquer diverses mesures urgentes pour lutter contre les fraudes sociales. À l’époque, cette proposition fut traitée comme marginale et considérée comme d’une efficacité non avérée. C’était pourtant mettre un pied dans la porte. Aujourd’hui, la lutte contre la fraude sociale est une cause majeure et unanimement partagée. Mes chers collègues, il me semble important de rappeler que cette proposition de loi n’est que le premier jalon d’une réforme nécessaire et attendue, qui se doit d’être bien plus vaste. Si ce texte se concentre sur certaines instances nationales, un effort similaire devra être engagé à l’échelon local. Plus globalement, globalement, il s’agira de poursuivre le travail des gouvernements successifs sur les agences et opérateurs de l’État. La commission d’enquête qui passera au crible dans les prochains mois le millier d’opérateurs et d’agences qui dépendent de l’État devra faire des coupes courageuses pour supprimer les doublons et les branches mortes. Rappelons également que plusieurs commissions et comités ne sont pas du ressort du législateur : leur nature réglementaire les place sous la seule responsabilité de l’exécutif, qui devra, lui aussi, amorcer un travail de rationalisation systématique. l’État et ses opérateurs, la Cour des comptes appelait le Gouvernement à s’interroger régulièrement sur la justification du recours à ce mode de gestion du service public. En conclusion, mes chers collègues, soutenir ce texte, c’est affirmer une volonté politique claire : celle de bâtir un État qui n’hésite pas à se réformer pour mieux fonctionner. Nous avons aujourd’hui la possibilité d’ouvrir la voie à une véritable réflexion de fond sur l’efficacité de l’action publique. Les sénateurs du groupe Union Centriste soutiendront, bien évidemment,

Face à la réduction croissante du nombre de fonctionnaires, aux enjeux nouveaux et au besoin d’accompagnement, de conseil et d’évaluation, de telles structures se sont, il est vrai, multipliées. Elles seraient désormais obsolètes, coûteuses et inutiles. Pourtant, c’est un débat beaucoup plus approfondi que nous devrions mener ici. Il ne s’agit pas de se cantonner à énumérer les comités qui doivent être supprimés. Ne donnons pas l’impression que l’objet de ces instances n’entre plus dans le champ des politiques publiques.

– Kanaky s’opposera toujours à la « casse » de l’État au nom de « l’efficacité gouvernementale », si chère au nouveau président outre Atlantique et à ses amis milliardaires, mais si néfaste pour notre société. L’efficacité d’un État, d’un comité, ne se mesure pas à court terme, mais s’évalue sur le temps long.

aucun impact sur les comptes publics, mais elle aurait des conséquences désastreuses sur le secteur. Nous prenons d’ailleurs acte des amendements visant à éviter cette suppression. garantit en effet les extensions d’accord à toutes les entreprises de la branche des industries électriques et gazières. Elle fait donc partie intégrante du statut, assurant ainsi un socle entre les agents. La supprimer serait une erreur. J’évoquerai également l’article 6, qui tend à supprimer la commission de suivi et de propositions de la convention visant à améliorer l’accès à l’emprunt et à l’assurance des personnes présentant un risque aggravé de santé. De nombreuses avancées ont été obtenues pour les personnes ayant un risque aggravé afin qu’elles puissent outrepasser les nombreuses difficultés pour accéder à l’emprunt. Les combats menés ne peuvent être balayés par notre empressement. Il semble donc que trop d’éléments aient été omis.

Cette commission est fondamentale pour l’indemnisation des victimes d’essais nucléaires. Le nombre de personnes potentiellement exposées aux retombées radioactives s’élève à 400 000 : 150 000 personnels civils et militaires ayant participé aux campagnes nucléaires, 210 000 Polynésiens et 40 000 Algériens.

Oui, il est nécessaire de supprimer les structures dépassées ou obsolètes. En revanche, il serait plus judicieux de ne pas rayer celles dont les enjeux sont si concrets en l’absence d’autres solutions. Qu’en est il, par exemple, de la commission nationale d’autorisation Aussi faible le nombre de demandes soit il, son existence répond à un vrai besoin de s’assurer des compétences des personnes qui seront en face de patients en attente de réponses sur des questions essentielles pour leur santé.

qui tranche parfois trop à l’aveugle dans des structures dont l’utilité est bien réelle. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission.

à Mme Nathalie Goulet. Il s’agit d’un amendement de Jean François Longeot. La Commission nationale d’aménagement commercial (Cnac) constitue une instance superflue dans la chaîne de décision relative aux projets d’aménagement commercial, alors même que les collectivités locales

Cela représente, pour l’année 2023, 181 saisines traitées, au cours de dix huit séances d’examen. Près d’une fois sur deux, l’autorisation initialement refusée est acceptée. Il s’agit donc d’une chambre d’appel extrêmement importante et fructueuse pour les élus locaux. Quel est l’avis du Gouvernement ? Pour les mêmes

Mme Nadia Sollogoub, pour explication de vote. C’est précisément pour cette raison que M. Longeot a déposé cet amendement : bien souvent, la décision départementale et la décision nationale ne vont pas dans le même sens.

Prévention et répression doivent s’articuler et, surtout, participer à l’évolution nécessaire des mentalités. L’individualisation des sanctions doit être également défendue, tout comme la fermeté des peines prononcées. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

sur le fond, ce comité, loin d’être inactif, joue un rôle essentiel dans la régulation des statistiques publiques et l’application du code des bonnes pratiques. Troisièmement, supprimer ce comité, ce n’est pas seulement supprimer une structure aussi supprimer des garanties essentielles, au premier rang desquelles l’obligation du secret statistique pour les bénéficiaires d’accès aux données. Est ce un risque que nous voulons réellement prendre ? Pour ces raisons, nous défendons activement le maintien de ce comité.

(CMT), instance directement rattachée aux services du Premier ministre et prévue par le législateur pour garantir la sécurisation des ordonnateurs dans le cadre des transactions financières les plus importantes. Son objectif principal est d’encourager le recours à la transaction, qui constitue un mode rapide et extrajuridictionnel de règlement des litiges. Chaque ministère est tenu d’instituer un CMT. Le comité ministériel de transaction présente un double intérêt. D’une part, il assure une instruction rigoureuse et approfondie, dans les domaines à la fois juridique et financier, des transactions portant sur des montants élevés. Ces dossiers donnent lieu à un avis écrit et signé. D’autre part, lorsque le signataire d’une transaction suit cet avis, sa responsabilité personnelle, à l’exclusion de la responsabilité pénale, ne peut être engagée.

de transaction en un comité interministériel unique. Néanmoins, cette fusion ne serait que purement cosmétique ! En effet, les transactions traitées étant spécifiques à chaque ministère, un tel regroupement n’améliorerait ni l’efficacité ni la pertinence des analyses effectuées. C’est pourquoi le Gouvernement vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, de bien vouloir entendre ses arguments

Nous avons là l’opportunité de passer de cinq instances consultatives à une, grâce à une mutualisation interministérielle qui me paraît de bon aloi.

du secteur, de la Confédération des grossistes de France et des distributeurs alimentaires spécialisés. Ils m’ont confirmé combien cette commission était utile et précieuse, parce qu’elle était un moyen de résoudre préventivement un certain nombre de de conflits commerciaux. De fait, cette commission, qui se réunit régulièrement, rend des avis et fait des analyses de jurisprudence, est un élément essentiel dans un paysage commercial qui, on en conviendra,

est un espace de travail qui, par l’engagement bénévole des associations qui y siègent, participe à faire avancer collectivement le développement de l’économie sociale et solidaire. Il s’apprête

d’une instance précieuse pour l’ensemble des acteurs de l’économie sociale et solidaire, pour la coconstruction des dispositifs et des politiques publiques prenant en compte les spécificités de ces entreprises. Ce conseil est organisé autour de nombreuses commissions, toutes actives.

qui incarne une autre forme d’économie, souhaitable et présente dans tous nos territoires. Quel

évidente. Toute politique publique n’a pas nécessairement besoin d’une instance de pilotage national ! Le pilotage peut être académique ou départemental.

Cette instance, qui existe depuis 2005, a pris différentes formes, a évolué dans sa composition, dans le nombre de ses membres, sans jamais véritablement faire ses preuves. Elle n’a d’ailleurs jamais réalisé la mission d’évaluation qui lui avait été confiée, ce qu’un rapport de l’inspection générale a souligné dès 2017. Elle ne s’est pas réunie

l’un dédié aux droits d’auteur, l’autre dédié aux droits voisins. Le collège « droits d’auteur » de cette commission est compétent pour faciliter la conclusion d’accords relatifs aux droits d’auteur des journalistes et, à défaut d’accord, fixer les modes et les bases de la rémunération due en contrepartie des droits d’exploitation. Le collège « droits voisins » de cette commission a pour mission de faciliter la conclusion d’accords relatifs au partage de la rémunération